monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues lors du jour appelle l'examen de 4 projets de loi tendant à autoriser la ratification l'approbation de conventions internationales pour ces 4 projets de loi, la conférence des présidents retenu la procédure d'examen simplifié, je vais donc les maîtres successivement aux voix. Pour la première, je mets au voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après un engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatives à des substances qui appauvrissent la couche de zones, la commission des affaires étrangères et favorable à l'adoption de ce texte donc sur ce texte qui est pour. Qui est contre, abstention donc le projet de loi est adopté. J'ai mis aux voix, le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération meurt, zone frontalière entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi frontalier d'aéronefs commission des Affaires étrangères et favorable à l'adoption de ce texte. Donc, qui pour corrompre. Pas d'abstention donc le projet de loi est adopté, je mets au voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement là. Procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcée entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part et la République du Kazakhstan, d'autre part, la commission des affaires étrangères et de la Défense et des forces armées et favorable à l'adoption de ce. Texte donc qui est pour qu'on ne trouve personne, pas d'abstention donc le projet de loi est adopté, dernière convention. Je mets au voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, sur la sécurité sociale, du 1er octobre 1980 relatifs aux soins de santé programmée dispensés en France aux ressortissants algériens, assurés sociaux et démunis non assurés sociaux, résidente en Algérie, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte, donc qui est pour. Contre personne pas l'abstention donc ce projet de loi est adopté. Donc, nous allons finir les l'ordre du jour appelle maintenant l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets plans et programmes et portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en l'absence du du rapporteur, je vais vous faire part des propos qui ne souhaitez-vous tenir ce matin, nous sommes en effet réunis ce matin pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 20 décembre en vue d'élaborer un texte commun sur le projet de loi ratifiant les ordonnances, numéro 2000 16058 et 2000 16060 du 6 août 2016 je ne reviendrai pas sur le contenu de ces 2 ordonnances dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter lors de l'examen du projet de loi en première lecture l'objectif principal est de moderniser plusieurs outils de procédure essentiel à la démocratie environnementale, qu'il s'agisse de la concertation préalable de l'évaluation environnementale ou de la participation du public au stade des procédures d'autorisation. La commission mixte paritaire a mené ses travaux dans un état d'esprit particulièrement ouvert et constructif, et je me félicite de l'accord que nous avons trouvé en bonne Intelligence avec l'Assemblée nationale en effet le texte élaboré par la commission mixte paritaire reprend des apports importants de chacune des 2 assemblées et constitue ainsi un compromis très équilibré concernant l'ordonnance relative à l'évaluation environnementale, le texte reprend 2 ajouts significatifs du Sénat qui correspondent à des propositions formulées dans le cadre du rapport de la commission d'enquête sur la compensation des atteintes à la biodiversité, dont le président était Jean-François Longeau et le rapporteur Ronan Dantec, le 1er rajout exige du maître d'ouvrage de répondent systématiquement par écrit aux observations formulées par l'autorité environnementale dans son avis rendu sur l'étude d'impact du projet qui fait l'objet d'une demande d'autorisation, l'objectif est court moment de la procédure de consultation du public tous les éléments, puisse être mis à disposition du public en toute transparence, cette disposition vise à conforter et à généraliser une pratique déjà fréquentes de la part des maîtres d'ouvrage. Le second apport reprend une proposition qui a pour but d'enrichir l'étude d'impact d'un projet par l'analyse de ses incidences sur la consommation d'espace agricole naturel, les forestiers, outre les effets du projet lui-même sa disposition intégrera l'impact sur le foncier des mesures d'évitement de réduction et de compensation, en effet, comme l'ont souligné les conclusions de la commission d'enquête, ces mesures peuvent elles-mêmes représentées des surfaces importantes qui s'ajoute à l'emprise des infrastructures elles-mêmes, il est important de prendre en compte l'ensemble de ces enjeux fonciers en vue d'améliorer l'insertion territoriale des projets concernant l'ordonnance relative à la participation du public le texte de la commission mixte paritaire reprend également plusieurs ajouts du Sénat à notre demande, a été en effet maintenu à 4 mois le délai dans lequel les vices de procédure ou de forme type de la participation préalables peuvent être invoquées par voie d'exception lors d'un recours contre la décision d'autorisation d'un projet, cela permettra de maîtriser les risques de contentieux et de conserver l'équilibre trouvé entre les différentes parties prenantes lors de l'élaboration des ordonnances par ailleurs, le texte reprend un ajout du Sénat visant à étendre aux collectivités territoriales, aux associations de protection de l'environnement, l'allongement à 4 mois du délai d'exercice du droit d'initiative que l'Assemblée nationale avait initialement réservé aux habitants, enfin l'Accord trouvé en CMP reprend une disposition que nous avions adopté en 1ère lecture en vue d'inscrire dans la loi une proposition de la mission commune d'information sur la démocratie de 2017 au collège Henri Cabanel et Philippe Bohn Carrère avaient été respectivement président et rapporteur, elle permet la désignation facultative d'un garant, chargé, chargé de la phase d'information et de participation, intermédiaire entre la concertation préalable en amont et l'enquête publique en aval pour les projets non soumis à la Commission nationale du débat public, l'objectif est d'améliorer la continuité de l'information et de la participation du public pour les différentes phases de réalisation d'un projet, au total, la commission mixte paritaire, a adopté un texte particulièrement équilibré et je me félicite que les discussions dans notre assemblée et permis de traduire concrètement plusieurs propositions formulées à l'issue de travaux de contrôle menée l'année dernière les 2 ordonnances enrichie par le Parlement, via le présent projet de loi permettront de renforcer la qualité environnementale des plans programmes et projets et d'en améliorer l'acceptabilité tout en proposant de réelles mesures de simplification pour les aménageurs, publics je vous invite donc à adopter sans réserve ce texte, je vous en remercie. donc, la parole est maintenant à monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire monsieur mini c'est à vous. Merci monsieur le président Monsieur, président de la commission du développement durable est mort et que le département de l'Eure occupe la tribune sur cette séance du matin qui a salué le rapporteur et l'ensemble des membres de la commission Alain Fouché, qui va nous rejoint, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me retrouver une nouvelle fois devant vous sur ces 2 ordonnances comme je l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale la semaine dernière, je suis particulièrement satisfait que collectivement nous soyons arrivés à à bâtir un texte particulièrement équilibré sur 2 ordonnances particulièrement technique, il faut bien le dire, l'une sur l'évaluation environnementale des projets plans et programmes et l'autre sur l'information à la participation du public lors de l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement tient plus particulièrement à remercier le rapporteur de la commission Alain Fouché pour le travail qu'il a menée sur ce texte depuis plusieurs mois et l'ensemble des parlementaires qui ont pris part à ce débat et, entre autres, vous Monsieur le Président Maurer votre démarche constructive, a permis d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire le 20 décembre dernier nous avons donc un texte issu de la CMP, qui est équilibrée, reprenant la majeure partie des dispositions adoptées à la affaire nationale et au Sénat, vous l'avez dit, monsieur le président, je crois que faire émerger un consensus sur un texte qui, précisément, traite de la concertation était important, je rappelle d'ailleurs que ces 2 ordonnances sont elle-même le fruit d'une concertation approfondie au sein de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique menée par le sénateur et ancien ministre de la Défense Alain Richard 2 ordonnances donc l'une relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets plans et programmes avec un objectif de simplification et de clarification des procédures, l'autre permettant de réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public avec une volonté d'associer davantage en amont les citoyens à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, bien entendu, c'est surtout la seconde ordonnance qui a donné lieu à d'importants débats entre les parlementaires et c'est bien normal car cette ordonnance était, je le rappelle, l'une des réponses du gouvernement de l'époque, un changement de mentalité dans notre société, qui s'est notamment opéré exprimé après le terrible drame de Sylvain j'aimerais rappeler 3, principale mesure de cette dernière ordonnance la première la création d'un droit d'initiative qui permettra au public, aux collectivités locales, aux associations de demander l'organisation d'une concertation préalable, en un mot de l'instruction d'un projet projet 2ème la mise en place d'une véritable concertation préalables en amont de l'instruction d'un projet plan au programme, nos concitoyens ont trop souvent pu avoir le sentiment que la participation intervenait trop tard pour leur permettent d'avoir une réelle influence sur le projet et sur le sens de la décision publique qui s'y attachent, préalables répond à cette critique et permettra d'apaiser localement les tensions qui peuvent parfois s'exprimer la 3ème avancée, c'est la soumission des plans programmes nationaux à une saisine de la commission nationale du débat public, connu sous l'acronyme de CNDP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, cela permettra d'associer le public pour des plans programmes encadrant la réalisation de projets le plus en amont possible au moment discussion sur les périmètres d'implantation de ces projets, c'est ordonnance a bien entendu des effets Directs et concrets souhaiterait prendre 2 exemples d'actualité pour illustrer la CNDP adorent, c'est déjà décidé d'organiser une première concertation préalables sur les documents stratégiques de façade, 4 grandes façades maritimes françaises qui a d'ailleurs déjà commencé, ce qui permettra de lancer un débat sur la planification spatiale de ces espaces maritimes et littoraux et bien sûr un 2ème débat public est cours il va démarrer bientôt au mois de mars sur la révision de la programmation pluriannuelle énergie la PPE et là aussi, le Parlement aura l'occasion, comme je vais déjà dit à de nombreuses reprises à cette tribune d'en connaître, je souhaite réaffirmer ici une conviction forte du gouvernement, la formation à la participation du public le plus en amont est un facteur de réussite de la transition écologique, porté par l'État et les différents opérateurs, je pense notamment au projet de méthaniseur ou d'éoliennes qui peuvent susciter, c'est légitime, parfois des inquiétudes, la concertation n'est pas une perte de temps, mais bien un moyen à la fois d'apaiser les tensions sur le terrain et de faciliter l'autorisation et la réalisation de ces projets dans des délais rapides, les sénateurs qui participeront participer au groupe de travail sur l'éolien et la méthanisation ont pu voir que la concertation est une priorité dans nos échanges, gage de premiers résultats, enfin j'aimerais rappeler les principaux points de consensus qui ont été émerger en commission mixte paritaire grâce à votre travail, premièrement la réintroduction d'un seuil maximal de 5 millions d'euros, dépenses publiques ou de subventions publiques, l'investissement pour déclencher le droit d'initiative, je sais que le Sénat, Monsieur le Président mourait étaient plutôt réticents à l'idée d'inscrire un seuil de 5 1000000 dans la Loire, rappelant que cela relevait davantage du réglementaire, alors que du côté de l'Assemblée nationale, cela constitue un marqueur important aussi, je tiens à vous remercier sincèrement et collectivement le rapporteur Alain Fouché, vous-même, Monsieur le Président, d'avoir accepté de réintroduire ce seuil dans un esprit bien connu ici au Sénat et que je salue le compromis car vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, l'ensemble des acteurs nous attendez et souhaite une ratification rapide de ces ordonnances le rapporteur à l'Assemblée nationale, le député Jean-Marc Tunisie a d'ailleurs adopté la même démarche sur un autre point en acceptant de conserver le délai de 4 mois fixé par le Sénat pour les recours en illégalité pour vice de forme deuxièmement, il a été réintroduit une articulation entre les procédures de concertation et débat public du code de l'environnement avec la concertation du code de l'urbanisme, les échanges en CMP ont permis d'aboutir à une rédaction répondant : je crois aux préoccupations des 2 assemblées, troisièmement, les parlementaires ont fait évoluer la rédaction d'une mesure introduite par le sénateur Ronan Dantec, si présent sur la prise en compte de la compensation écologique sur la consommation d'espace agricole dans les études d'impact des projets, les débats ont été nourris en CMP sur ce sujet après plusieurs échanges vous êtes parvenus là aussi une rédaction de compromis et je m'en félicite le gouvernement présentera tout à l'heure un amendement purement rédactionnel sur ce point, en accord avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, à des fins de qualité d'écriture de la loi, mais là, messieurs les sénateurs, comme j'avais pu le dire en première lecture, apprendre à perdre du temps en amont d'un projet ou d'une procédure est nécessaire pour ne pas en perdre ensuite consulter plus largement nos concitoyens permettra de lever les doutes qui peuvent parfois exister sur certains projets, il est désormais urgent de ratifier ces ordonnances nationale veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évaluation sur leurs effets, je me suis engagé devant vous et je le redis ce matin à la tribune du Sénat je réaffirme moment engagement d'avoir une évaluation rapide de leur application, le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance des sacs que vous allez prochainement examiné prévoit justement un rapport sur l'ordonnance, information et participation du public, un délai de 2 ans pour produire son rapport me paraît raisonnable pour évaluer les premiers effets de l'ordonnance en attendant, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président, Monsieur le président de la commission, je vous propose de doter ce texte issu de la CMP, fruit de l'excellent travail que vous avez su mener c'était mon baptême du feu sur mon 1er texte en tant que membre du gouvernement je tiens donc à vous en remercier. Merci monsieur le ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nelly Tocqueville. Non, Monsieur le président, Monsieur le ministre Monsieur le président de la commission du développement durable, ce mais, chers collègues, je tiens à préciser donc si la Normandie qui est présente jusque-là lors de l'examen, donc en première lecture de ce projet de loi ratifiant 2 ordonnances du 3 août 2016 relatives à l'environnement j'avais souligné le caractère consensuel et transpartisan de ce texte je me satisfait donc du succès de la commission mixte paritaire du 20 décembre dernier, rappelons que l'article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron habilite le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, notamment dans le domaine du droit de l'environnement, au total 6 ordonnances auront été prises sur la base de cet article en comptant les 2 présents, je l'avais signalé le 10 octobre dernier, celles-ci vont dans le bon sens l'initiative du précédent gouvernement, dans la rédaction de ces ordonnances doit une nouvelle fois être salué, ainsi que les longs mois de travaux qui ont abouti à un large consensus avec les différents acteurs, ce projet de loi s'inscrit donc pleinement dans le principe de continuité républicaine, auquel nous sommes tous attachés pour rappel dès 2014 suite à la conférence environnementale, plusieurs groupes de travail se sont réunis cette riche concertation les travaux menés en lien avec la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique présidée par notre collègue Alain Richard ont permis cette modernisation du droit de l'environnement, à l'issue de ce travail, un rapport a été rendu par les présidents des groupes de travail, Jacques Vernier, en mars 2015, les ordonnances s'en inspire, nous l'avions précisé très largement celle-ci comme il a été souvent rappelé sont en quelque sorte une réponse au drame du barrage de Sylvain et aux événements dramatiques que nous connaissons ces ordonnances sont d'autant plus essentiel qu'elle repose tout d'abord sur les grands principes, notamment l'article 7 de la charte de l'environnement, laquelle, rappelons-le, a valeur constitutionnelle et consacre le principe du dialogue environnemental aussi a le réaffirme le principe figurant dans la loi de la reconquête de la biodiversité, à savoir la séquence éviter réduire compenser pour mémoire la première ordonnances portent sur la réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur nos vies, rendement, la 2ème est relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets plans et programmes ainsi instauré à haut niveau de dialogue et de participation du public ainsi qu'une nécessaire qualités environnementales sont des objectifs primordiaux que nous nous devons de développer et de de promouvoir sans détailler l'ensemble des dispositions proposées par ce projet de loi, je tiens à souligner quelques mesures phares qui témoigne de la volonté d'atteindre ses objectifs fait ici référence au renforcement du rôle et des prérogatives de la Commission nationale du débat public à la création d'un droit d'initiative citoyenne pour l'organisation de concertation préalable à certains projets au renforcement de la transparence et à la famille facilitation de la participation du public à la concertation, notamment par une plus grande dématérialisation ou enfin la clarification des procédures d'évaluation environnementale pour les projets, plans et programmes comme j'ai pu le dire lors de l'examen en première lecture ce projet de loi est d'autant plus important qu'il permet de transposer la directive européenne relative à l'évaluation environnementale des projets et d'améliorer la conforme du doigt français au droit de l'Union européenne et de sa cour de justice, en cela, nous répondons donc à l'exigence de mise en conformité et nous ne pouvons que nous en satisfaire les modifications survenues en commission mixte paritaire me semble là aussi répondre à cette volonté de travailler ensemble des compromis, vous l'avez rappelé ont été trouvés sur la majorité des points de divergence, et ce dans l'intérêt de tous, je me félicite particulièrement que cette CMP et retenu le seuil de 5 millions d'euros à partir duquel le nouveau droit d'initiative citoyenne pour l'organisation d'une concertation préalable sur certains projets peut-être activé et que j'avais défendue par voie d'amendement enfin ces textes permettent des simplifications, sans pour autant réduire l'exigence de protection de l'environnement, c'est pourquoi le groupe socialiste et républicain du Sénat, est satisfait de cet accord trouvé entre les 2 chambres dans cette commission mixte paritaire et votera donc, par conséquent, ce texte, toutefois, soyons conscients qu'il reste encore beaucoup de travail à effectuer sur ces sujets et qui sera certainement nécessaire dans les prochains mois, d'évaluer l'efficacité de ces ordonnances et ProB probablement d'améliorer certains points comme vous venez de le préciser, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci donc

il est temps qu'un Breton prennent la parole, sinon ça semblait commence à ressembler à l'hémicycle normaux, monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de vin. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les 2 ordonnances qui nous est aujourd'hui proposé de ratifier s'inscrivent donc cela a été dit dans ce long chantier de modernisation du droit de l'environnement, qui s'est engagé sous la précédente mandature, nous sommes je crois tous favorables au fait chercher à faire progresser l'évaluation environnementale et la participation du public dans les procédures conditions incontournables à des débats apaisée, nous sommes tous conscients, je crois, des difficultés dans la conduite des projets en France à travers l'actualité régulière démobilisation, voire des affrontements qui ont accompagné utilise maintenant le passé certains grands projets d'aménagement avec des risques réels sur l'a été rappelé le drame du mais aussi à travers les blocages dénoncé constamment de colloque en colloque, par exemple sur le développement de de l'éolien, il y a donc aujourd'hui, je crois, un intérêt commun entre les grands aménageurs, les associations de protection de l'environnement pour trouver des réponses au blocage par des processus d'évaluation globale des projets et des débats publics transparent où toutes les données sont maintenant vraiment sur la table sur ce point particulier, l'éolien, je tiens d'ailleurs à souligner l'engagement du ministre sur cette question sur la simplification des installations d'éoliennes, c'est un des vrais facteurs de retard de la France aujourd'hui dans la transition énergétique et c'était un chantier ex-absolument essentiel, je tiens, moi aussi à souligner, cela a été dit l'important travail de concertation réalisé en amont du texte discuté aujourd'hui dans le cas des groupes de travail présidée par le sénateur Alain Richard et aussi par Jacques Vernier insisterai sur 2 points précis de ces ordonnances qui me semble particulièrement important énorme et novateur l'ordonnance sur l'évaluation environnementale complet le contenu de l'étude d'impact et souligne tout particulièrement, cela n'a pas été redit l'introduction dans cette analyse de l'incidence du projet sur le climat et sur sa vulnérabilité face aux dérèglements climatiques, cela devrait aussi nous amener à évaluer donc demain, certains grands projets d'infrastructures de transport au regard de leurs émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, l'étude d'impact se fait également plus précis sur la biodiversité, il faut désarmer décrire les mesures envisagées pour respecter la séquence éviter réduire compenser et définir plus précisément, point important, le suivi des mesures compensatoires, ce qui constitue une avancée dans le sens de la loi pour la reconquête de la biodiversité et des préconisations de la commission d'enquête du Sénat sur ces compensations des atteintes à la biodiversité dont j'étais donc le rapporteur, comme l'a rappelé le président donc je ne peux être évidemment que satisfait de l'adoption définitive de nos 2 amendements qui se baser sur les conclusions de cette commission d'enquête, que présidait Jean-François longs jours je tiens aussi à noter à souligner le caractère fructueux des échanges qu'on a eue avec nos collègues de l'Assemblée nationale sur ce point en CMP n'est-ce pas Alain Fouché et je crois qu'ils ont été sensibles à nos argumentaires comme vous la aviez était monsieur le ministre, en séance ici au Sénat, même si après on n'a pas senti un enthousiasme complet de l'état et qu'il a donc fallu rester mobilisés, donc le 1er de ces amendements tend à revenir sur l'impact de se poser sur l'agriculture notamment sur ce point aujourd'hui essentiel de la consommation du foncier agricole en oubliant donc pas d'analyser non seulement la consommation de foncier liées aux infrastructures, mais aussi la impact en terme de mesures compensatoires donc avoir une vision beaucoup plus globale de l'impact sur l'économie agricole, l'autre amendement adopté définitivement rendons systématique la réponse écrits du maître d'ouvrage sur la vie de l'autorité pour éviter que les les comptes Estacion naturaliste ne surviennent après l'enquête publique, le fait que l'avis de l'Autorité environnementale sont maintenant complétés par cette réponse écrite du maître d'ouvrage, à des éventuelles objections doit permettre un débat plus approfondie et donc aussi plus apaisé, c'est un point important de nature à réduire les contestations qui interviennent souvent il faut le rappeler après l'enquête publique elle-même au cours de laquelle donc tous les sujets n'ont pas été abordés, notamment au moment des arrêtés de la loi sur l'eau, il s'agissait d'une conclusion importante de la commission d'enquête au Sénat je suis évidemment très heureuse que ce soit maintenant dans la loi, nous n'avons pas issu Monsieur le Ministre, mais je sais que vous en partager la préoccupation sur cette fameuse clause filer ou clause de de rattrapage la rédaction actuelle nous semble toujours fragile car les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise que tout projet impactant sérieusement l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, mais donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra revenir les ordonnances ne répondront pas à tous, mais les exigences de transparence, de dialogue, de contre-expertise d'approche globale des projets sont au coeur d'un débat public apaisée dont nous avons tous besoin, aujourd'hui, l'État est maître d'ouvrage se sont souvent montrés frileux, méfiant sur ces débats en pensant que, finalement, plus donner d'informations, plus il nourrissait la contestation notre analyse est inversé la faiblesse du débat qui nourrit aussi les contestations, nous pouvons donc souligner les avancées progressives qui sont intervenues ces dernières années et l'accord qui me semble assez consensuel sur le texte et donc un signal positif supplémentaire si j'étais un cas, je dirais même un 2ème signal positif apportée par l'État et la représentation nationale sur une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et, en 1er lieu de biodiversité dans les projets d'infrastructures, le groupe RDSE votera donc évidemment les conclusions de la CNP, je dis simplement, peut-être en conclusion, je pense que Nelly Tocqueville dit aussi un petit peu, on a aussi devant nous tout un processus de simplification administrative, il faudra être extrêmement vigilant dans ce cadre de simplification, on ne revienne pas en arrière par rapport à tout le travail qui a été menée pour un débat apaisé sur les enjeux environnementaux, je vous remercie. Merci monsieur Dantec donc la parole est maintenant à monsieur Guillaume Chevron liés.

je vais pas lui vanter un vain suspense le groupe Les républicains votera bien sûr pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables le Sion environnemental et portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public une telle issue était rendue possible par le travail de notre rapporteur Alain Fouché, qui dès la première et unique lecture a travaillé avec un vrai esprit de synthèse et, encore une fois, la majorité sénatoriale s'est se montrer constructive, monsieur le Ministre dans ce projet de loi, il n'a échappé à personne que l'enjeu ne portait pas sur la ratification des 2 ordonnances précitée, personne ne peut en effet s'opposer à une réforme qui doit permettre de simplifier la vie quotidienne des collectivités territoriales et des professionnels, tout en assurant une meilleure implication de nos concitoyens, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, lors de la l'examen du projet de loi en première lecture la première ordonnance répond à la nécessité de simplifier le parcours des maîtres d'ouvrages en prévoyant une étude d'impact par projet et non plus par procédure tous les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés y sont favorables, la nécessité de soumettre pour avis le document d'évaluation environnementale avant autorisation du projet à la consultation des collectivités territoriales, fait l'unanimité. S'agissant de la seconde ordonnance avec le renforcement de la concertation en amont et processus d'autorisation et ensuite la modernisation de la concertation en aval, là encore, aucune difficulté. Pour notre groupe politique, l'enjeu de cette commission mixte paritaire résidait dans les 3 points cardinaux suivant l'inscription dans la loi d'un seuil à 5 millions d'euros de dépenses prévisionnelles pour un projet afin de permettre l'accès à un droit d'initiative du public 2ème point le passé de 4 à 6 mois le délai durant lequel l'illégalité pour vice de forme ou de procédure peut-être invoquée par voie d'exception 3ème point allongé A4 au lieu de 2 le délai offert pour exercer un droit d'initiative citoyenne en ce qui concerne la suppression de l'allongement à 6 mois du délai durant lequel l'illégalité pour vice de forme ou de procédure peut-être invoquée, c'est la position du Sénat qui l'a emporté, s'agissant de l'allongement à 4 mois du délai offert pour exercer un droit d'initiative citoyen la position de sagesse du rapporteur consistant à étendre cet allongement à l'ensemble des parties prenantes, y compris aux collectivités territoriales, était la seule solution envisageable je rappelle ici qu'il fallait harmoniser ces délais pour la recevabilité de la demande d'autorisation à l'expiration du délai d'exercice du droit d'initiative, le plus long, soit 4 mois je me réjouis que la voix exprimées par le Sénat était entendu, même s'il s'agissait de considérations effectivement très technique, dernier point cardinal de l'examen en commission mixte paritaire le seuil des dépenses prévisionnelles pour un projet afin de permettre l'accès à un droit d'initiative du public sur ce sujet la position défendue par la majorité sénatoriale n'a pas été comprise en effet c'est ajout nous semble contraire à l'article 41 de la Constitution car les manifestement de rang réglementaire au final sur les 3 sujets majeurs qui restaient en discussion à l'examen de la commission mixte paritaire issue ont été ont trouvé une issue favorable à la position exprimée par le Sénat, le dernier point étant beaucoup plus politique, on ne pouvait pas discuter à armes égales avec la majorité de l'Assemblée nationale pour cette raison et parce que le projet de loi est guidée par la volonté d'alléger les contraintes administratives pesant sur les collectivités territoriales et sur les professionnels, notre groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire et et comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, espérons que ce texte permettra de favoriser la réalisation de projets de méthanisation de projets photovoltaïques permettant ainsi à notre pays d'être pleinement dans la transition énergétique, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole maintenant à Madame Éliane Assassi. Monsieur le président Monsieur ministre, chers collègues, la Seine-Saint-Denis s'intéresse aussi à tous ces sujets, contrairement à ce que certains pourraient penser donc ce texte, nous l'avons examiné ce texte qui ratifie 2 ordonnances du 3 août 2016, nous l'avons examiné en première lecture au tout début du mois d'octobre, c'est-à-dire 2 semaines après les élections sénatoriales, les délais extrêmement courts n'avait pas à leur permis un travail approfondi sur un texte particulièrement technique, puisque ce sont 60 articles du code de l'environnement, qui ont été créés ou modifiés, la CMP s'est tenue donc en décembre dernier dans une ambiance constructive et un texte de compromis a été adopté à l'unanimité sur les 2 articles restant en discussion, nous en prenons acte, même si nous estimons que certaines dispositions instaurées par le Sénat auraient dû être supprimés CMP, il en est ainsi de l'instauration d'un délai de 4 mois pour soulever un vice de forme dans une procédure dure au titre de la concertation, le délai fixé à 6 mois à l'Assemblée par l'Assemblée, nous sommes satisfaits que la CMP et restaurer un plafonnement du seuil de dépenses publiques à partir duquel un projet et soumis à déclaration d'intention et un droit d'initiative ce seuil étant fixé à 5 millions le Sénat avait fait le choix de ne pas fixer ce seuil, renvoyant à la prise d'un décret, ce qui nous semblait constituer une incompétence négative du législateur à la fin du processus législatif, nous continuons de nous interroger sur certaines dispositions contenues dans ses ordonnances et sur la méthode utilisée, nous regrettons ainsi mais vous le savez, le recours à la pratique des ordonnances, conjugué à la déclaration d'urgence qui prive les parlementaires de leurs prérogatives législatives, les réduisant à un simple contrôle à posteriori de dispositions déjà intégrées déjà intégrées dans le droit positif, or cette méthode de gouvernement et de plus en plus utilisé pour aboutir aux dispositions les plus efficace et pertinente le travail parlementaire a besoin de temps, il ne s'agit pas là de temps perdu, mais bien du temps nécessaire de formation de la décision publique dans une démocratie, sur le fond, alors que l'exigence d'une meilleure association du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement tant à s'exprimer, de plus en plus fortement au sein de la société, nous regrettons que l'ordonnance ne soit pas à la hauteur ni des enjeux ni des attentes, soyons clairs, si l'objectif est d'éviter pour demain des drames comme celui de Siemens, rien ne nous permet aujourd'hui de dire que ces dispositions portent le début du commencement de réponse en effet au-delà des reformulation clarification et nouvelles compétences confiées à la Commission nationale du débat public plutôt positive en terme de concertations préalables, le droit d'initiative créé reste très encadrée, ce qui nous fait craindre l'émergence d'un droit purement fictif, ouvrir un droit nouveau, en plaçant des conditions matérielles inatteignable pour sa mise en oeuvre est de nature à générer une frustration inutile et donc il semble donc une démarche contreproductive dans ce cadre, nous partageons les regrets de notre collègue, Barbara Pompili, président de la commission du développement durable de l'Assemblée, qui a alerté la commission mixte paritaire et le gouvernement sur la difficulté à de réunir 500000 citoyens pour saisir la commission nationale du débat public sur un projet de réforme de politique publique telle que le prévoit l'ordonnance que nous devons ratifié je rappelle alors que nous avions porté un amendement sur le sujet, permettant de diviser par 2 ce seuil sans que celui-ci ne reçoivent un avis positif ni du gouvernement ni de la majorité sénatoriale même sort pour notre proposition de rendent plus efficient, le droit d'initiative citoyenne pour les projets de plus faible ampleur en transformant le contrôle d'opportunité du préfet en une simple formalité pour constater constater que les mêmes conditions matérielles formulée par la loi soient remplies, au final, ce droit d'initiative des corrélée à aucune obligation de prise en compte par le maître d'ouvrage qui l'affaiblit considérablement permettent l'expression est une chose, encore faut-il que cette expression puisse être entendus, il serait alors opportun de prévoir une évaluation de la mise en oeuvre réelle de ces dispositifs après l'entrée en vigueur de la présente loi pour vérifier si, comme nous le craignions il s'avère peu opérationnel sur l'ordonnance relative aux évaluations, nous avons depuis le début de l'examen de ce texte, une vision extrêmement critique de ces dispositifs, qui passe d'une évaluation environnementale systématique à une évaluation au cas par cas, selon l'appréciation des services de l'État, or la faiblesse des moyens, notamment humains dans les directions régionales de l'environnement, de l'Aménagement et du logement, laisse craindre d'un contrôle minima a minima, ce qui n'est malheureusement pas nouveau en matière de respect de l'environnement, nous regrettons enfin l'absence comme nous l'avions proposé avec le sénateur Dantec d'une cloche, il en a parlé, pour éviter que des projets petits par leur dimension mais un fort impact environnemental puissent faire l'objet d'une évaluation pourtant l'arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2017 impose au gouvernement de mettre fin à la possibilité d'une régression du droit en matière de protection de l'environnement, le gouvernement aurait pu. Proposé lors de la CMP, une proposition en ce sens afin de respecter le droit européen et la jurisprudence administrative, elle aurait été acceptée, me semble-t-il, pas nos assemblées, malheureusement, cette question a été renvoyée vers un autre véhicule législatif et pour l'ensemble de ses réseaux, nous confirmons donc notre vote défavorable de la première lecture. Chers collègues, merci, donc, la parole est maintenant monsieur Philippe bonne. Oui,

Oui, monsieur le président, Monsieur le secrétaire d'État mais, chers collègues, les 2 ordonnances qui nous sont soumises cultive les bonnes intentions, a salué par définition, c'est le temps et l'expérience qui nous en donnerons il il faut me semble-t-il laisser vivre cette réforme dans la globalité des 4 ordonnances pour apprécier, par exemple, si d'autorisation environnementale unique sera en pratique un succès fondamentalement je crois que les textes qui nous sont soumis, relève d'une transition, ils partent à juste titre de l'idée que la manière de décider a changé dans notre société, nos concitoyens aspirent à s'exprimer de manière concrète et continue sur un croissant de sujets et donc de nombreux domaines de l'action publique, l'environnement n'y fait pas exception le développement de cette démocratie environnementale repose en partie sur l'affirmation des droits, l'information et à la participation du public droits nouveaux qui doivent être concilié avec la nécessaire poursuite des projets d'infrastructures pour les promoteurs du texte protection de l'environnement, participation du public et faisabilité des infrastructures ne sont pas antinomiques, l'objectif est d'associer davantage nos concitoyens, j'ai indiqué à la prise de décisions dans le domaine environnemental tout en permettant au maître d'ouvrage de mener à bien leur projet, c'était un exercice de curseurs seront de régulation auquel nous sommes conviés je n'écarte pas, mais les points de vue peuvent être différents et nous venons de l'entendre en écoutant Madame que le balancier souhaite aller un peu trop loin à la défaveur de la capacité à faire et à faire de manière qualitative à l'aube de ses objectifs, les ordonnances que nous sommes sur le point de ratifier porte sur de nombreux sujets, des avancées et je tiens à remercier l'ensemble des collectes pour le travail constructif accompli en particulier monsieur rapporte parmi les accords de compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire plusieurs mérite d'être salué concernant l'ordonnance relative à la participation du public, l'abaissement de 6 à 4 mois du délai pour les recours en illégalité pour vice de forme ou de procédure rééquilibre un peu le texte, je me réjouis également que des conclusions de la mission d'information sénatoriale sur la démocratie participative ou coopérateurs que j'ai partagé avec l'un de nos collègues de de l'Hérault était intégrée au texte de l'ordonnance en particulier la désignation facultatif dans garant, chargé de la phase d'information et de participation intermédiaire, j'insiste sur l'intérêt d'expérimenter une procédure continue monsieur d'une ministre de consultation du public, la désignation d'un grand sur le temps long permettra d'assurer la transparence et la médiation tout en favorisant le bon déroulement du projet et j'ai vu que dans divers textes, vous commencez à en intégrer certains éléments, je pense aussi aux propositions que nous avions pu faire sur le fait de respecter le double degré de juridiction tout en commençant certains domaines par un recours devant la cour d'appeler administratif avant bien sûr la possibilité de saisir le Conseil d'État, enfin, je tenais à saluer l'pour choix opéré par la commission mixte paritaire d'opter pour une logique de simplification une convergence entre les règles du code de l'environnement et celle du code de l'organisme, alors que l'Assemblée nationale avait décidé de privilégier la concertation du code de l'environnement à celle prévue par le code d'urbanisme, nous avions au contraire fait le choix d'une convergence des 2 codes afin de réduire les délais des opérations tout un assurant un niveau de garantie similaire, si l'accord de compromis qui a finalement été trouvé diffère quelque peu puisque la concertation au type du code de l'environnement primera toujours, du moins dans 5 sont montrés dans une approche trop technique, il n'en demeure pas moins qu'une étape a été franchie en terme de lisibilité des procédures, le Sénat auraient apprécié monsieur ministre que sinon la fusion du moins, la coordination des 2 côtés de l'environnement et de l'urbanisme soit privilégiée, globalement, mais notre collègue Alain Richard qui va me suivre à cette tribune, Anne avait déjà mesuré la difficulté lorsqu'il avait travaillé sur le rapport qui a été largement un un point toutefois suscite en nous une certaine inquiétude, le fait d'avoir privilégié la voie législative pour la fixation du seuil à partir duquel les projets relèveront du droit à l'initiative, il avait pourtant été admis que cette disposition avait intrinsèquement une nature réglementaire et que son encadrement par la loi et réduirait toute future adaptabilité du soleil, faute d'accord entre donnent aux assemblées, l'Inde des décidé autrement, mais ce choix n'est pas de nature à changer notre regard sur ce texte mais, chers collègues, le groupe de l'Union centriste, votera le texte proposé par la commission mixte paritaire dont nous partageons, sinon la lettre, du moins l'esprit, il est peut-être un peu sévère comme j'ai entendu il y a quelques secondes ou quelques minutes de dire qu'il n'y avait pas dans ces dispositions, le début du commencement d'une d'une réponse Madame Assassi peut-être de manière un petit peu différente, qu'il y a bien sûr une part de risque dans les ordonnances, proposer, du moins dans leur mise Anna, par contre je crois profondément, avec mes collègues qu'il y aurait un risque plus emportant aujourd'hui à ne pas donner une place importante à la dimension participative dans la réalisation de projet ou dans la dimension environnementale au sens large, je terminerai en indiquant que la notion de transition me paraît cependant assez présent et que le caractère transitoire de ces dispositions nous conduira y revenir sinon court terme je pense qu'il faudrait mieux l'éviter du mois au moyen terme et si vous en doutiez, chers collègues, Lady régime dérogatoire que vous avez voté la semaine dernière en votre présence, monsieur le ministre, au sein du texte consacré aux jeux olympiques ensemble annonce la confirmation, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur, bonne Carrère, la parole est maintenant Madame Colette Mélot.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mais, chers collègues, la commission mixte paritaire des rapporteurs Alain Fouché, que je salue tout particulièrement mon cher collègue et Jean-Luc Jules les il est parvenu à un compromis, à quelques jours des fêtes de fin d'année 2017, nous pouvons nous en féliciter, débuté en avril 2017 l'étude du projet de loi de ratification des 2 ordonnances du 3 août 2016 a connu une histoire mouvementée, déposée par l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal retiré en juin 2017 puis redéposé par le nouveau ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, il a été adopté par l'Assemblée nationale dès le mois de juillet mais a parallèlement été modifié par le Sénat. Pour en comprendre les enjeux, il faut remonter plus loin encore dans le temps, l'article 106 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron prévoyait que le gouvernement soit habilité à réformer par ordonnances les règles applicables à l'évaluation environnementale en réformant ses procédures relatives au projet Plan ou programme affectant l'environnement, la loi vise à mieux associer le public aux décisions et à lui assurer une plus grande transparence sur la décision publique à nous 2016, le gouvernement avait donc pris 2 ordonnances relatives à ces questions d'évaluation environnementale l'ordonnance numéro 2000 16058 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale opère un 1er revirement stratégique elle fait passer le droit d'une évaluation systématique à une évaluation au cas par cas pour concentrer nos forces sur les projets ayant le plus d'impact sur l'environnement, l'ordonnance de 1016 1060 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public renforce la concertation un amont du processus décisionnel, elle propose de nouveaux outils, élargissement du Champ du débat public aux plans et programmes, création d'un droit d'initiative citoyenne ou encore attribution de nouvelles compétences à la Commission nationale du débat public complété par 2 décrets d'application, d'août 2016 et d'avril 2017 ces ordonnances ne sont pas seulement une avancée en droit français, elles sont aussi un impératif de mise en conformité avec le droit européen, il me semble ainsi utile de rappeler que la France avait avait avait eu un peu l'objet en mars 2015, d'un avis motivé de la Commission européenne, jugeant incomplète et fermer la liste des plans et programmes soumis à des vols valu à Sion il y a donc un véritable enjeu à traduire le droit européen dans les plus brefs délais pour éviter d'éventuelles sanctions administratives et financières ces ordonnances, mes chers collègues, modernise notre façon de considérer la vie du citoyen dans le processus décisionnel, plus que jamais notre droit doit donner une information parfaite et compréhensible à chaque citoyen et lui permettre d'exprimer une opinion sur les grands projets en renforçant la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et plan ces ordonnances nous permettent donc d'aller de l'avant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire : Sébastien Lecornu. Assurer les Hummer en une formule simple : l'enjeu majeur de ce projet de loi, il faut apprendre à perdre du temps Anne d'un projet pour ne pas le perdre, ensuite en simplifiant et clarifiant les règles un améliorant l'articulation entre les évaluations et le lancement des projets en renforçant enfin la concertation ces ordonnances nourrissent une révolution des pratiques de notre pays, monsieur le président, Monsieur le ministre mais, chers collègues, le groupe les indépendants républiques et territoires soucieux d'être à l'écoute de la parole citoyenne favorable aux 9 initiative de débat public votera en faveur du texte issu de la CMP, convaincu de sa capacité à changer la donne, nous lui accordons toute notre confiance et espérons qu'il puisse véritablement nous aider à franchir une prochaine étape dans l'aménagement de notre territoire vous remercie. Madame Mellow merci donc la parole est maintenant à monsieur Alain Richard. C'est le président Monsieur Miss, mes chers collègues, les textes dont nous allons ratifier l'adoption par ordonnance et qui sont déjà en vigueur, poursuivait en réalité 2 objectifs principaux : le 1er concernant l'évaluation environnementale était de concentrer l'effort de cette évaluation et la charge procédural qu'elle implique sur les projets les plus importants, les plus significatifs et le second d'instaurer familiariser dans notre public, un système de participation préalables en début de projet le moins formaliste possible pour faciliter les rapprochements de points de vue entre les citoyens et les porteurs de projets. C'est déjà une satisfaction dans l'action publique, de dire que une partie de ses objectifs. En ce qui concerne la concentration sur les projets essentiels. De l'évaluation environnementale, il y a juste un obstacle mineur auquel on est bien obligé de se référer, qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne, monsieur le ministre vous le Découvrez ignore l'interministériel

donc ce produit assez fréquemment que des directives ou des règlements soit adopté, avec un seul angle de vision de l'intérêt général européen et c'est le cas de beaucoup de directives en matière environnementale, qui considère que l'environnement suivant une expression qu'on a entendu sur d'autres sujets, ça n'a pas de prix et donc ça n'a pas d'impact financier et économique de compétitivité, etc, et donc les règles de l'Union européenne, auquel nous avons souscrit sans doute avec un peu de légèreté exclut tout seul en matière de besoins l'évaluation environnementale, adopté une schéma de compromis que nous faisons fonctionner tant bien que mal avec le système du cas par cas on ce que consolider ce que restreint un peu dans la mesure du raisonnable l'ordonnance que nous allons finir d'adopter par la ratification, c'est un système qui présente des obstacles qui présentent des difficultés pour les praticiens, puisque le cas par cas et lui-même conçu consommateur de Guinée et facteur d'incertitude mais nous ne ferons pas mieux, sauf à faire un jour une une révision de des pratiques souhaitée par l'Union européenne en ce qui concerne la participation préalable, en revanche, là, nous sommes parvenus parce qu'on était dans un espace un peu plus de liberté à la concentrer sur les projets à la réguler, disons la concentrer sur les projets les plus susceptibles de donner lieu à des désaccords et en arrivant en parvenant à mettre à l'abri, l'essentiel des projets entrepreneuriaux puisque globalement, seuls les projets émanant de collectivités publiques bénéficiant de de financements publics substantiels sont assujetties à cette démarche de concertation près préalables et lorsque il m'a été demandé, avec un groupe représentatif de dire organisation du CNT de réfléchir à ce sujet, on était arrivé au diagnostic que malgré parfois des impact réel sur le terrain, la plupart des projets d'autorisation d'établissements classés sont ceux qui sont portés par les entreprises représentent une très faible minorité dans les projets réellement controversé, donc il y a un système de prévention à la à la à la main des préfets qui me semble-t-il, répond indiquent-ils donc. Au terme de cette évolution lève l'allégement relative de l'évaluation et la clarification directe de l'évaluation environnementale est un acquis qui est au moins satisfaisant, a salué et la concertation préalable commence prendre disons son son démarrage et il faudra apprécier si elle permet, en effet, des approches coopérative des approches qui permettent de rapprocher les points de vue de la représentation des citoyens et les porteurs de projets, ou si au contraire elle joue le rôle, simplement d'une anticipation des oppositions et les blocages, auquel cas il faudrait en prendre conscience, lors de l'évaluation qui sera nécessaire une dernière observation, nous finissons en février 2018 un processus. Auxquels il était demandé une certaine rapidité à la fin 2009, de moi qui suis un des rares soldats perdus dans les assemblées parlementaires à défendre les ordonnances parce que je crois que, de temps en temps, c'est une bonne façon de faire avancer les textes, je dois reconnaître que d'être passée par des ordonnances pour mener le travail en 3 ans et demi ne va pas énormément dans le sens de mon plaidoyer alors il y a eu entre-temps une alternance qui, c'est vrai, a retardé la à retarder l'approbation la le processus de ratification mais entre le lancement du processus d'ordonnances et l'adoption des ordonnances, il s'est écoulé un délai qui aurait pu être raccourcie, parce que lorsque le gouvernement ne délibère avec lui-même et avec ses conseils, ça prend parfois presque autant de temps que le temps du débat parlementaire, donc je ne rend pas les armes, je continue à penser que les ordonnances peuvent rendre bien des services à une législation de qualité, encore faut-il en avoir la détermination merci. Monsieur Richard merci donc la discussion générale est Close, je rappelle qu'en application de l'article 42 alignés à 12 du règlement, le Sénat examinant après Assemblée Nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou accepté par le gouvernement, donc nous passons à la présentation des amendements du gouvernement. Donc premier amendement sur l'article de Monsieur le Ministre, l'actionnaire je crois. Oui, monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs je si vous m'y autorisez monsieur le président, une présentation commune des 2 amendements qui, comme je l'ai dit, lors de la discussion sont des amendements de porter rédactionnel pour revenir juste ajuster les choses suite à la CNP. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur, sur les 2 sur les 2 amendements qui sont sur l'article 2 sur l'article 5. Merci Monsieur le Président, simplement 2 mois auparavant, merci, même l'Lambesc et de ce retard est dû à un incident important indépendant de la volonté, je sais que le président Maurer du chose excellemment, donc je n'ai pas de soucis, je voudrais dire aussi que je me félicite que du travail qui a été réalisé entre nos 2 assemblées sur la qualité des débats et du travail qui a été réalisée aussi avec le ministre, donc avec le gouvernement, je le projet de loi traduit bien à la fois le respect de l'environnement tout en apportant souplesse modernité simplification, ce qui en définitive amènera à plus d'efficacité sur ces 2 amendements, c'est un avis favorable. du texte élaboré par la commission modifié par les amendements du gouvernement il y a-t-il des explications de vote. Non, c'est un vote bloqué amendement et était de la

à nouveau me me réjouir de cet accord que nous avons trouvé en CMP, ça a été largement dit je, je n'y reviens pas, je crois que c'est un bon accord qui prend en compte les points de vue des 2 assemblées et notamment les positions de notre haute assemblée et j'en profite pour dire au gouvernement que cela montre que nous sommes prêts à travailler à la fois avec l'Assemblée nationale et aussi avec le gouvernement, et si je dis ça, c'est pas totalement par hasard c'est parce que ces derniers temps, nous avons eu le sentiment que lorsqu'un texte venait du Sénat, il était par principe jugé par l'assemblée par le gouvernement comme un mauvais texte, nous avons vécu cela avec la proposition de loi du président Retailleau sur l'assainissement qui, arrivé à l'Assemblée nationale a tout de suite été renvoyé en commission alors que dans le même temps, les députés de la majorité, sortez un texte qui s'inspirait très fortement de cette proposition de loi, nous n'avons vécu la semaine dernière lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue pas rapporter excellemment par Didier Mandelli sur la question du du Toral ou la secrétaire d'État brune Poirson, n'a pas voulu entrer dans la discussion n'a pas voulu amender le texte considérant que, bien sûr, il y avait pas, il y avait pas lieu à l'et on a appris peu après qu'en fait, le cabinet du ministre d'État préparait, je cite, une proposition de loi et loi et bien entendu le gouvernement prépare une proposition de loi qui sera porté par des députés, et pas plus tard qu'hier, nous avons auditionné en commission, le secrétaire d'État au numérique Julien Normandie que nous avons interrogé sur la suite que le gouvernement entendait donner à la proposition de loi que nous examinerons début mars de de notre collègue Patrick Chess destiné à sécuriser les réseaux d'initiative publique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été assez on va le sort ou la suite que le gouvernement entendait réserver à cette proposition doit donc si ça Monsieur le Ministre, c'est pour que vous entendiez vous fassiez passer le message à l'ensemble du gouvernement, le fait que c'est pas parce qu'un texte vient du Sénat, que c'est un mauvais texte et que le Sénat n'est nullement dans une posture politicienne dans une plus dure d'opposition, nous sommes prêts à fortiori sur des sur des sujets comme cela qui dépasse largement les clivages politiques à travailler en bonne entente avec l'Assemblée nationale et le gouvernement, je remercie. Merci monsieur Maurer, il n'y a pas d'autre explication de vote. Non, donc je mets aux voix à l'ensemble du projet de loi. Dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire modifié par les amendements du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre l'abstention. Donc le projet de loi est définitivement adoptée, je vais suspende la séance, elle sera reprise à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est suspendue.